J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de la commission des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête afin de mener une mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance d'hier, mercredi 19 janvier.

affaires sociales. En conséquence, la commission des affaires sociales se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission d'information. Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d'être prise par le Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier. J'invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières.

Cet accord traduit l'objectif partagé par nos deux assemblées de donner aux acteurs de la protection de l'enfance des outils destinés à mieux protéger et accueillir les enfants en danger. Grâce au travail parlementaire, le texte du Gouvernement se trouve enrichi de dispositifs qui permettront de répondre aux attentes et aux besoins des professionnels et des enfants. Je vous invite donc à adopter ce texte, qui comporte de nombreux dispositifs approuvés ou ajoutés par le Sénat. Tout d'abord, ce texte permettra d'accueillir les mineurs protégés dans de meilleures conditions et de renforcer la prévention des risques de maltraitance dans leur prise en charge. Sur l'initiative du Sénat, l'accueil de mineurs protégés dans des hôtels sera totalement interdit d'ici à deux ans. a précisé que, dans l'intervalle, cet accueil ne pourrait se faire pour plus de deux mois et qu'il serait encadré. Cette mesure ambitieuse et nécessaire pour la protection des enfants représente une avancée majeure pour laquelle les départements devront se mobiliser dès la promulgation de la loi.

pour autoriser l'exercice d'une activité dans le secteur social ; les antécédents judiciaires des personnes vivant dans l'entourage des assistants familiaux et maternels La prévention des risques de maltraitance sera mieux formalisée dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; ceux-ci se doteront d'un référent indépendant qui pourra répondre aux difficultés des personnes accueillies. La mise en place d'une base nationale répertoriant les agréments des assistants familiaux, étendue par le Sénat aux assistants maternels, donnera aux départements une visibilité sur les retraits et les suspensions d'agrément prononcés dans d'autres territoires. Le texte complète et ajuste les modalités d'accompagnement et de prise en charge des mineurs protégés, pour mieux s'adapter à leurs besoins et favoriser leur autonomie. L'Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi approuvé, dès la première lecture, la nécessité d'étudier systématiquement la possibilité de recourir à un tiers digne de confiance, de proposer à l'enfant d'être accompagné par un parrain, de faciliter la désignation d'un avocat pour l'enfant, de permettre le recours à une médiation familiale, ou encore de mettre en place des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée. L'accompagnement jusqu'à 21 ans des jeunes en difficulté sera systématique. Le Sénat a en outre introduit la possibilité d'un droit au retour pour ceux qui se sont éloignés de l'aide sociale à l'enfance, mais souhaiteraient être de nouveau soutenus par les départements. Rappelons, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement s'est engagé à accompagner financièrement les départements pour assurer la prise en charge effective de ces jeunes en difficulté. Les conditions de travail des assistants familiaux seront améliorées : leur rémunération sera au moins égale au SMIC, ils pourront bénéficier de week-ends de repos et participeront davantage aux décisions importantes concernant l'enfant. Ces dispositions, certes utiles, ne seront toutefois pas suffisantes pour enrayer le déclin démographique de cette profession. Concernant la protection maternelle et infantile (PMI), nous avons, avec nos collègues députés, adopté un dispositif équilibré, qui permettra de concilier une logique d'objectifs d'activité et la garantie de normes minimales d'effectifs pour les services de PMI, dont les actions d'accompagnement des familles sont essentielles pour la prévention des risques de maltraitance et de carences éducatives. Enfin, la gouvernance de la protection de l'enfance, qui souffre aujourd'hui de cloisonnements et d'hétérogénéité, Les instances nationales de la protection de l'enfance devraient ainsi se regrouper au sein d'un seul groupement d'intérêt public (GIP). Ce regroupement, approuvé par le Sénat, permettra d'harmoniser les pratiques professionnelles par la collecte d'informations et la diffusion de référentiels. par la commission mixte paritaire reprend également les dispositions introduites par le Sénat, qui visent à améliorer la coordination de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance sur le terrain et à prévenir les ruptures de parcours des enfants. À cette fin, nous avons proposé d'instituer des comités départementaux de la protection de l'enfance, coprésidés par le président du département et le préfet, afin que l'ensemble des acteurs se réunissent et coordonnent leur action. Leur institution, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, est la condition de leur succès et de leur appropriation par les départements. Il nous reviendra ensuite collectivement, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de veiller à l'appropriation et à l'application effective des mesures de ce projet de loi. Je vous propose donc d'adopter ce texte qui, dans le prolongement des lois de 2007 et de 2016, offre aux collectivités et aux professionnels des outils pour mieux protéger les enfants et améliorer leur prise en charge. La parole est à M. le secrétaire

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, cher Bernard Bonne, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que l'examen de ce projet de loi relatif à la protection des enfants touche à sa fin, me reviennent en mémoire les mots, les visages, les joies et les peines exprimées par les centaines, sans doute même les milliers d'enfants que j'ai eu la chance de rencontrer depuis trois ans, depuis que j'exerce mes fonctions au sein du Gouvernement. Certains d'entre eux ont eu des existences cabossées, des parcours compliqués, mais toutes et tous partagent le même souhait, la même aspiration : grandir sans crainte ni appréhension, s'épanouir dans un quotidien fait des mêmes chances, des mêmes droits et des mêmes opportunités, bref, être des enfants comme les autres, ni plus ni moins. On dit souvent que le poste que j'occupe a été créé en réponse à la diffusion de documentaires et d'enquêtes dévoilant la face sombre de notre système de protection de l'enfance. C'est faux dès 2018, avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Président de la République avait mis l'enfance au coeur de la lutte contre les inégalités de destin. Ce secrétariat d'État en était le prolongement naturel et nécessaire.

et, demain, à son application, en passant bien sûr par la démarche de contractualisation pluriannuelle entre l'État et les départements, fondée sur des objectifs partagés et des moyens financiers dédiés, la dynamique engagée a été construite sur la base de la responsabilité partagée. Je pense que seul un travail collaboratif entre l'État, les départements, les associations, les professionnels et les enfants est source d'améliorations durables de la situation de ces derniers. J'ai mené ce travail en repartant des fondements des précédentes lois relatives à la protection de l'enfance, celles de Philippe Bas et de Laurence Rossignol, que je salue. Les acquis de ces lois font aujourd'hui consensus ; ils auront été, à divers égards, des points de repère dans ma démarche de ces derniers mois.

Dernière traduction de cette méthode, j'avais très tôt annoncé mon souhait de laisser ce texte ouvert, de laisser la version présentée en conseil des ministres s'enrichir des apports du Parlement.

Ce texte doit marquer la fin d'une époque faite d'incertitudes et d'insécurité pour ces enfants, à qui nous garantissons un cadre de vie sécurisant et serein, et pour les adultes qu'ils deviendront. par l'Assemblée nationale, des mesures fortes avaient été retenues, introduites par les députés, mais également par le Gouvernement. Je pense ainsi à la mesure prévoyant, à l'article 1, d'étudier systématiquement la possibilité de confier l'enfant à un tiers digne de confiance, accompagné et soutenu,

en fonction du parcours qu'il souhaite construire, de ses attentes et de ses envies pour sa vie future. Je pense enfin à la valorisation de la parole de l'enfant. Auditionné systématiquement en tête-à-tête par un juge des enfants, il pourra désormais être bien plus régulièrement représenté ou défendu par un avocat ou un administrateur.

Placées sous le signe de l'intérêt des enfants, qui nous aura tous guidés au cours de nos débats, elles auront contribué à transformer en profondeur la protection de l'enfance. Je salue ainsi les mesures concrètes prises pour assurer au quotidien la sécurité des enfants.

même si l'on peut toujours souhaiter que cela aille plus vite et plus loin. Je souhaite que cette expérimentation puisse se déployer dans les meilleurs délais ; j'appelle à cette occasion les départements à faire acte de candidature pour que le plus grand nombre d'entre eux rejoignent cette démarche favorisant, me

Cette réforme, complémentaire des 100 millions d'euros que l'État a remis en trois ans à la PMI, au travers de la contractualisation avec les départements, permettra de pérenniser cette politique fondamentale à laquelle nous sommes tous attachés.

État, département, secteur associatif habilité, société civile doivent être éclairés sur l'impact des politiques suivies, sur les évolutions quantitatives et qualitatives des besoins, sur les perspectives à retenir ». C'est tout l'objet de cette réforme, d'apparence technique, mais dont l'objectif est bien de renforcer notre expertise commune sur ces sujets et de renforcer le pilotage de la protection de l'enfance dans notre pays, au bénéfice des enfants et des professionnels. De la même façon, nous travaillerons au déploiement rapide de la base nationale des agréments pour les assistants maternels et familiaux. Par ailleurs, d'ici quelques mois, l'extension de la vérification des antécédents judiciaires des personnes travaillant au contact d'enfants sera effective, ce qui garantira qu'aucune personne ayant été condamnée, notamment pour des infractions sexuelles, ne pourra intervenir auprès d'eux.

qui sont actuellement protégés et les personnes qui l'ont été à un moment de leur vie, pour les échanges que nous avons eus. Avec ce texte, nous posons la dernière brique de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance d'octobre 2019. Même s'il restera toujours à faire pour encore mieux protéger nos enfants à l'avenir, nous pouvons déjà être fiers de cette étape. Nous passons

Qu'une loi de protection des enfants intègre des dispositions relatives à la gestion des flux migratoires n'est pas tolérable ! L'obligation faite aux conseils départementaux de consulter et de renseigner

ils y voient les prémices de la fin des institutions, des foyers et des maisons d'enfants à caractère social (MECS). D'autres, dans le secteur de la pédopsychiatrie, dont on connaît la situation actuelle, craignent les conséquences psychologiques de cette

tu ou excusé les souffrances, s'ils sont dignes de la confiance que la société leur confère pour protéger l'enfant de sa famille toxique. Cette disposition permettra-t-elle d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux des enfants et, en premier lieu, de leur méta-besoin de sécurité ?

Il s'agit d'une compétence partagée, exercée entre l'État et les départements, aux côtés des institutions scolaires, judiciaires et sanitaires. La tentative d'expérimenter un comité local annuel me fait l'effet d'une parodie de gouvernance, comme si l'on hésitait entre la recentralisation prônée par certains et la mise sous tutelle de collectivités manquant d'ambition pour la protection des enfants.

Le contrôle des antécédents de violences sexuelles de l'ensemble des personnes au contact des enfants mérite également d'être salué, comme l'attention accrue portée aux fratries Enfin, notre groupe se félicite d'avoir permis d'adosser au SMIC la rémunération des assistants familiaux, dans une démarche de revalorisation d'un métier en mal d'avenir.

Nous nous abstiendrons donc, en regrettant que ce rare temps législatif accordé à la protection des enfants aboutisse à si peu. La parole

la commission mixte paritaire, réunie le 11 janvier dernier, a trouvé un accord sur le projet de loi relatif à la protection des enfants. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de la discussion générale en première lecture, ce texte comporte de belles avancées. ces belles avancées figure l'accueil prioritaire des fratries dans un même lieu. Nous savons en effet le déchirement que peut provoquer une séparation pour des frères et soeurs qui partagent des liens affectifs souvent forts et une histoire commune.

sera enfin un outil efficace pour protéger davantage les enfants, où qu'ils se trouvent. L'amélioration des conditions d'exercice du métier d'assistant familial a été au coeur de nos débats. Cette profession fait face à de nombreuses difficultés auxquelles nous devrons répondre, puisque 40 % des assistants familiaux partiront à la retraite dans les quatre prochaines années. une tâche immense, puisqu'ils participent pleinement à la reconstruction des enfants placés, dont le parcours est souvent chaotique. La question de la revalorisation et de l'attractivité de leur métier devra faire l'objet d'une attention toute particulière dans les mois et les années à venir, si nous voulons qu'ils continuent à remplir leur mission dans les meilleures conditions.

me semble disproportionné, tout d'abord, au regard de l'intérêt de l'enfant, supérieur à toute autre considération. En effet, le temps de l'enfant n'est pas celui de l'adulte. Deux ans, dans la vie d'un enfant, c'est une éternité ! En outre, disons-le,

Les départements qui ont recours à l'hébergement hôtelier ont donc déjà eu plus d'un an et demi pour adapter leur mode d'accueil. Leur laisser un an de plus à partir de la promulgation de la loi pour y mettre fin et organiser la transition vers d'autres modes d'hébergement plus protecteurs des enfants nous semblait donc raisonnable.

En tout état de cause, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi, qui apporte des réponses concrètes. Je crois néanmoins essentiel de repenser notre système de protection de l'enfance en profondeur durant les mois et les années à venir. Les disparités entre les territoires demeurent trop importantes et causent une rupture d'égalité entre des enfants qui bénéficient de politiques ambitieuses et protectrices et d'autres, qui n'ont pas cette chance et sont victimes de choix budgétaires contestables. je fais miens les propos du Président de la République prononcés devant les maires de France : il indiquait, à juste titre, que les Français ne votaient pas pour cent politiques différentes de protection de l'enfance ou du handicap. Je partage ce constat, car, quand il y a des dysfonctionnements dans les départements- et il y en a -, c'est vers l'État que l'on se tourne. C'est donc à lui de reprendre la main afin de rétablir cette égalité de traitement et de garantir à chaque enfant une protection digne sur l'ensemble du territoire. Ce projet de loi permettra de concrétiser de belles avancées afin d'améliorer le quotidien des enfants sous protection et leur accompagnement vers l'autonomie. Il constitue ainsi une étape importante dans la réflexion que nous devrons mener en faveur d'une meilleure harmonisation des pratiques et d'une protection digne des enfants placés.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, réformer en profondeur la protection des enfants était essentiel, même si des améliorations ont été recherchées au fil des années et que des évolutions seront toujours nécessaires tant le sujet est d'importance. Comme l'a déclaré Barack Obama, « ceci est notre première tâche : prendre soin de nos enfants ». La protection des enfants doit rester une attention de tous les jours. Protéger et accompagner les plus fragiles doit être une priorité. Depuis quelque temps, le Gouvernement promettait un texte à la hauteur des enjeux. Nos débats dans cet hémicycle, s'ils ont démontré le caractère crucial des propositions, ont mis en lumière les espoirs et les volontés. Le constat le plus frappant portait sur les différences de situations, parfois très larges, en fonction des territoires. Je salue les efforts qui ont été accomplis afin de garantir une uniformité dans la protection des enfants. avant d'en venir plus précisément aux avancées marquantes de ce texte, laissez-moi revenir une nouvelle fois sur deux points que j'ai évoqués lors de l'examen du texte en première lecture. Le premier, c'est le voeu que j'ai formé de voir la création d'un ministère régalien de l'enfance et de la jeunesse. L'objectif est simple : la clarification, l'unification de la politique dans ce domaine central. Le second concerne le harcèlement en ligne. Vous connaissez mon engagement sur ce sujet. Les violences numériques dont les enfants sont victimes sont en augmentation et sont de plus en plus importantes. Leur protection est cruciale.

Donnons-lui des armes pour mieux utiliser ces outils, mais aussi des moyens de se défendre et se protéger. Je suis optimiste : la prise de conscience a eu lieu, nous devons désormais offrir des solutions répondant à ces enjeux.

les jeunes sont livrés à eux-mêmes sans accompagnement adéquat, ce qui n'est pas acceptable. Il faut aider les acteurs de la protection de l'enfance en leur donnant les moyens de recourir le moins possible à cette pratique. Je salue donc le travail de réécriture de l'article 3. Grâce

Je le rappelle, la société entière doit se saisir de la protection de notre jeunesse. Sur ce point précis, je reste persuadée que la multiplication des mentorats entre les étudiants des grandes écoles- pourquoi pas aussi des facultés

Je trouve que l'attention qui a été portée à la gouvernance, notamment territoriale, va dans le bon sens. Le fait de réunir les acteurs, pour assurer le bien-être des enfants et l'efficacité des décisions prises les concernant, est une avancée notable. Accompagner nos jeunes et protéger les plus vulnérables d'entre eux est un engagement de chaque instant. Le fait que les liens entre les acteurs soient resserrés devrait être bénéfique à la fois pour leur travail et pour le quotidien des enfants. la commission mixte paritaire nous paraissent la solution à nombre de problématiques rencontrées dans le cadre de la protection des enfants. Il en reste malheureusement encore bien d'autres. C'est pourquoi nous continuerons inlassablement de travailler pour le bien-être de nos enfants, pour contribuer à leur épanouissement et assurer leur avenir, qui est aussi le nôtre.

l'objectif de ce projet de loi devait nous rassembler, tant les enfants qu'il concerne connaissent de difficultés. Ce fut le cas, malgré un certain nombre de divergences. La protection que nous devons à ces enfants est en effet au coeur de nos valeurs républicaines.

Il était important de se montrer pragmatique et de lutter, par exemple, contre les sorties précipitées de l'aide sociale à l'enfance. Ce droit au retour, pour les jeunes majeurs ayant quitté toute prise en charge, est crucial afin d'éviter toutes formes de décrochage, que nous savons dévastateur pour ces jeunes adultes. mes chers collègues, je ne reprendrai pas toutes les mesures ! -, nous avons souhaité éviter qu'un parent qui s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale ne la retrouve en cas de décès du parent l'exerçant. Vous l'imaginez bien- l'actualité nous y aide malheureusement parfois -, ce n'est pas un détail et il faut se réjouir qu'un accord ait pu être trouvé

Le personnel exerçant dans le champ social et médico-social est la pierre angulaire de cette politique publique. Je tiens ici à leur exprimer toute ma reconnaissance. est un véritable sacerdoce et je regrette que ce projet de loi ne prévoie pas une réelle revalorisation de ces professionnels, sur qui reposent tant de responsabilités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons adopté des dispositions qui sécurisent leur rémunération.

Ce dernier précise que ces contrôles devront s'appuyer sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Toujours dans le but de mieux protéger ces enfants, l'inscription dans ce fichier de toute personne vivant au domicile des assistants familiaux et maternels, y compris les mineurs de plus de 13 ans, fera obstacle à la délivrance d'un agrément.

Afin d'en assurer un pilotage efficace dans les départements, il a donc été prévu, à titre expérimental, une instance de pilotage partagé entre le président du conseil départemental et le préfet.

Ce dernier interdit l'hébergement des jeunes de l'ASE dans des hôtels, et ce dans un délai de deux ans. Afin d'inciter les départements à abandonner ce mode d'hébergement,

D'autres mesures concernant les mineurs non accompagnés ont été acceptées, notamment celles qui visent à renforcer leur accompagnement lors de l'entretien réalisé avant leur majorité. Précisons que, toujours pour éviter des décrochages, ce texte crée un nouvel entretien six mois après leur sortie de l'ASE. Aussi, mes chers collègues, il faut se féliciter que les deux assemblées se soient accordées sur la révision de la répartition territoriale des MNA, mais aussi sur l'interdiction des réévaluations de la minorité- oui, enfin ! -et sur le recours au fichier d'appui à l'évaluation de cette minorité Certes, ce texte n'est pas la grande loi attendue, ni même celle qui était promise, mais, pour ces enfants, il est important d'avoir pu avancer en bonne intelligence.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous nous retrouvons de nouveau autour d'un projet de loi qui ne met pas un terme à la politique en demi-teintes qui caractérise la protection de l'enfance, dans les moyens alloués sinon dans les objectifs affichés. relative à la protection de l'enfant, ce texte manque singulièrement de souffle. Certes, le travail parlementaire a étoffé ou conforté le texte de mesures positives texte de mesures positives comme l'instauration d'un droit au retour pour les jeunes majeurs, l'accompagnement des MNA dans leur demande de titre de séjour, la systématisation du parrainage, le renforcement du droit pour l'enfant à un avocat, la non-séparation des fratries et la valorisation des assistants familiaux.

la somme de ces dispositions ne suffit pas à définir une politique systémique en capacité de répondre aux problèmes structurels et récurrents de la protection de l'enfance, aggravés par une insuffisance de moyens, de places, de personnels qualifiés, malgré l'implication des équipes éducatives, sociales et médicales. La question est bien celle-ci : ce texte est-il à la hauteur des constats ?

Les autres enfants ou jeunes adultes décohabitent de chez leurs parents en moyenne à 25 ans et trouvent leur premier emploi à 22 ans. Remplissons-nous pareillement notre rôle de suppléance parentale ce texte de fin de mandat avance sur les sorties sèches, mais très- très -insuffisamment. Il faut faire beaucoup plus et aider les départements pour mettre fin à cette inégalité de destin, d'autant que les mesures de la loi de 1996, je pense aux projets pour l'enfant, sont très insuffisamment appliquées. dans son discours du 6 janvier dernier devant la Fédération des acteurs de la solidarité, a déclaré que, malgré ce texte, nous ne pouvons pas dire que nous ayons mis fin au déterminisme social qui frappe les jeunes sortant de l'ASE. Pour cela, il conviendra aussi de faire participer davantage les enfants et leurs associations aux décisions et orientations. Nous avons sans succès proposé des amendements en ce sens. Enfin, les mesures positives sont percutées

Il a été impossible de revenir sur certaines dispositions les concernant, obsolètes et indignes, comme les tests osseux. Nous déplorons non seulement la généralisation du fichier AEM, qui répond à des considérations largement étrangères à l'objet de ce le refus de respecter le principe de présomption de minorité et les droits de protection qui en découlent. Ainsi, si le texte apporte des améliorations dont il reste marqué par son manque d'ambition, qui est en partie dû au refus d'y consacrer de réels moyens. Une ancienne campagne du Secours populaire français pour les vingt ans de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) avait des droits de l'enfant (CIDE) avait pour slogan : « Les droits de l'enfant grandissent les hommes ». Force est de constater que, malgré ces avancées, le texte du Gouvernement nous empêche de bien grandir.

du côté des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance tout d'abord, qui aspirent à un statut social et à un accompagnement jusqu'à l'âge de 25 ans ; attentes du côté des personnels de la protection de l'enfance, des professionnels des centres de protection maternelle infantile et des centres médico-psycho-pédagogiques, des acteurs de la justice des mineurs ensuite, qui, tous, revendiquent des moyens supplémentaires et une revalorisation de leurs métiers. Face à autant d'attentes, il était sans doute difficile de satisfaire tout le monde, mais, faute de répondre à l'ensemble des revendications, tous resteront L'accord trouvé en commission mixte paritaire sur les quarante-trois articles restant en discussion permet des progrès. Je pense notamment au renforcement des contrôles des antécédents judiciaires du personnel social et médico-social, à la revalorisation des rémunérations des assistants familiaux, à l'attribution prioritaire d'un logement social aux mineurs de l'ASE ou à la possibilité de désigner un avocat pour les enfants capables de discernement.

mais c'est bien peu au bout du compte. Le 3 janvier dernier, vous avez participé à l'inauguration de la nouvelle maison départementale de l'enfance de Cergy, qui accueillera soixante-dix enfants. Ce nouveau site a nécessité un investissement de 13 millions d'euros.

nous voyons clairement l'écart considérable entre les arbitrages de Bercy et la réalité des besoins. Une autre question concerne vos propositions pour lutter contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Plutôt que de garantir l'accès aux contrats jeunes majeurs à tous les jeunes majeurs de moins de 21 ans, le Gouvernement préfère étendre des dispositifs d'aide qui ne sont pas adaptés. Pour notre part, nous sommes favorables à la création d'un statut social pour les jeunes majeurs de 18 à 25 ans. Nous regrettons également que l'article 2 relatif à l'autorité parentale en cas de violence ait été supprimé.

par le maintien dans le texte de dispositions qui sont sans rapport avec la protection des enfants, mais qui concernent plutôt la politique migratoire. Nous maintenons notre opposition aux tests osseux pour évaluer la minorité des enfants et le fichage automatique des enfants par les départements. Cette confusion entre politique migratoire, protection des enfants et contrôle de l'ordre public porte préjudice à l'image de la France, terre d'asile et d'immigration.

L'Assemblée nationale a amendé le texte, en particulier sous l'impulsion de Perrine Goulet, députée de la Nièvre, qui a grandi dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance et qui a fait de cette cause l'un des moteurs de son engagement. Les mesures élaborées ont visé à assurer un socle commun de droits pour tous les enfants, à soutenir tous les professionnels et à assurer une meilleure coordination entre tous les intervenants. Le Sénat, en commission et en séance, a poursuivi le débat en gardant pour guide un principe de réalité, celui des moyens des conseils départementaux, qui sont au coeur de l'action. Je souligne le travail remarquable de Bernard Bonne, rapporteur, qui, par son expérience d'élu, a une excellente connaissance du dossier. Il a fait preuve, lors de l'élaboration de son rapport et de ses propositions, d'une humanité et d'une capacité d'écoute que je tiens à souligner et dont je tiens à le remercier très sincèrement. La commission mixte paritaire a permis de finaliser certains points qui ont fait consensus, en particulier le versement à la famille de l'allocation de rentrée scolaire uniquement lorsque l'enfant réside au domicile d'un membre de sa famille, la sécurisation et l'anticipation de l'accès à l'autonomie des jeunes ne bénéficiant ni de revenus ni de soutien familial, la prise en compte des jeunes qui se livrent à la prostitution comme des victimes devant relever de mesures de protection, la possibilité pour le président du conseil départemental de saisir le bâtonnier en vue de la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et d'un administrateur pour l'enfant non capable de discernement, les conditions de mise en oeuvre du week-end de repos mensuel introduit pour les assistants familiaux.

plusieurs dispositions législatives du champ de la protection de l'enfance n'étant actuellement pas encore mises en oeuvre, comme sur celui de faire une nouvelle usine à gaz, qui ne règle ni les disparités territoriales ni les aberrations administratives.

nous comptons sur vous pour que ce texte, que vous avez défendu, vive dans les foyers de l'ASE, dans les familles d'accueil, dans les parcours de ces petits cabossés. Je termine mon propos en citant un grand homme, d'abord parce qu'il est nivernais, ensuite parce qu'il est assistant familial dans une petite commune rurale. Il a livré son témoignage dans la presse locale Depuis que je suis assistant maternel, je sais pourquoi je me lève le matin. Pour faire ce métier, il faut deux choses : avoir un grand coeur et être cinglé. » Nous lui devons bien cela, à lui qui essaie chaque jour de réparer des enfants amochés.

Cette dynamique, qui s'inscrit dans un cheminement législatif entamé à la fin du XIX siècle, nous conduit aujourd'hui à examiner un texte qui, selon notre groupe, permettra une meilleure prise en compte des besoins de l'enfant. Nous saluons donc le travail accompli en bonne intelligence par la commission mixte paritaire. L'une des avancées majeures de ce projet de loi est l'interdiction totale d'héberger des mineurs dans des hôtels. Nous connaissons les limites et dangers de ce dispositif : les mineurs y sont proches des lieux de trafic et les éducateurs trop peu présents.

En attendant, je ne peux que saluer la limite d'accueil de deux mois introduite par la commission mixte paritaire. Je me satisfais également qu'un pan de ce texte soit consacré à l'amélioration des garanties procédurales pour l'enfant en matière d'assistance éducative. notamment la désignation par le juge d'un avocat pour l'enfant capable de discernement. Je m'interroge cependant sur certaines notions que signifie être capable de discernement ? Être mature ? Avoir conscience de sa propre volonté ? Être responsable ? Le droit à être entendu est un droit fondamental, qui ne peut être conditionné à ces définitions encore trop obscures. Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d'exprimer à sa manière son bien-être ou son mal-être, en présence de la personne pressentie pour l'accueillir.

bon augure. Ces derniers, en effet, sont bien souvent confrontés à la réalité violente de la protection des enfants, enfants qu'il faut savoir accueillir et transformer sans tressaillir. L'équilibre psychique et la santé mentale des professionnels intervenant auprès des enfants ne peuvent donc être négligés. Malgré toutes les avancées concrètes recensées, je ne peux m'empêcher de revenir sur les silences de ce projet de loi, sans pour autant remettre en cause son bien-fondé. Une fois encore, je regrette que la question du suivi psychologique des enfants placés ne soit pas abordée. Il est inconcevable que des enfants témoignant d'une histoire difficile, souvent violente, ne soient pas suivis en bonne et due forme. Il est primordial de faciliter des processus de reconstruction psychique, lesquels restent encore trop chaotiques.

je suis choqué des propos indignes qui ont été tenus sur l'article 1. Je suis le ministre qui s'est le plus engagé contre l'inceste, et ce depuis très longtemps. Je me suis exprimé sur ce sujet. Aussi, dire que l'article 1

de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (texte de

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire (CMP), réunie le 14 décembre dernier, est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, autrement appelées thérapies de conversion. conversion. L'accord a été obtenu assez rapidement, la commission mixte paritaire ayant retenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, le texte que le Sénat avait adopté. En première lecture, le Sénat a notamment cherché à apaiser les craintes que la proposition de loi avait pu susciter sur l'accompagnement des personnes transgenres, en précisant qu'une invitation à la prudence et à la réflexion avant d'engager un parcours de transition ne saurait évidemment tomber sous le coup de la loi. Nous avons également complété le texte sur le sujet de l'autorité parentale afin que le juge pénal se pose la question, en cas de condamnation d'un parent, Nous avons ajouté, enfin, une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par un médecin et que la victime est mineure. Ces modifications ont enrichi la proposition de loi sans remettre en cause ses objectifs il s'agit de sanctionner des pratiques d'un autre âge qui prétendent modifier, des pseudo-thérapies ou des rituels religieux, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Si ces pratiques semblent, heureusement, peu répandues dans notre pays, il me semble important que la représentation nationale pose un interdit clair dans le code pénal, lequel exprime les valeurs et les principes auxquels une société est attachée. Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire, afin que ce texte puisse entrer rapidement Notre vote marquera l'aboutissement d'un travail de réflexion et de conviction entamé il y a déjà plusieurs années, sur l'initiative, notamment, de la députée Laurence Vanceunebrock. a d'abord conduit une mission d'information, avant de déposer la présente proposition de loi, dont elle fut rapporteure à l'Assemblée nationale. Je sais que nous pourrons ensuite compter sur l'engagement des acteurs du monde judiciaire et sur la mobilisation du monde associatif pour faire vivre ces nouvelles dispositions sur le terrain. Au-delà de cet aspect répressif, il nous faut poursuivre inlassablement un travail de pédagogie et d'éducation, notamment auprès des jeunes générations, afin de continuer à faire reculer les discriminations et les préjugés dont sont victimes les personnes homosexuelles ou transgenres. La parole est à Mme

madame la rapporteure- chère Dominique Vérien -, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, tout le sens de notre engagement politique est de rendre possible ce qui est souhaitable.

Les thérapies de conversion n'ont pas lieu d'être dans notre pays. Elles sont l'antithèse de nos valeurs républicaines d'égalité, de liberté et de fraternité. Non, on ne choisit pas son orientation sexuelle. Non, on ne choisit pas son identité de genre. Non, il n'y a rien à guérir. Et non, être soi n'est pas un crime ! Pendant trop longtemps, les souffrances engendrées par ces pseudo-thérapies ont été tues.

C'est pourquoi je me réjouis que la commission mixte paritaire soit rapidement parvenue à un accord sur ce texte, qui est un pas supplémentaire sur le chemin de l'égalité pour les personnes lesbiennes, gays,

électrochocs. Il est vrai que certains aspects de ces prétendues thérapies de conversion peuvent déjà être sanctionnés par un ensemble de dispositifs figurant dans le code pénal. Mais nous devions aller plus loin. La création d'un délit spécifique était nécessaire parce que ces agressions étaient méconnues. D'aucuns en ignoraient, voire en minimisaient la violence. Et si certains en doutaient encore, l'actualité nous a rappelé en début d'année cette réalité crue. L'histoire d'Enzo, cet adolescent transgenre envoyé contre son gré dans un établissement où sont pratiquées des thérapies de conversion, illustre la nécessité du texte qui nous réunit. Le Gouvernement a immédiatement saisi le procureur de la République sur cette affaire. Ce texte suscitera une prise de conscience collective sur l'ampleur et la gravité de tels comportements. Il permettra aux victimes de passer plus facilement la porte des commissariats pour briser le silence et l'omerta. Il mettra les forces de l'ordre et les magistrats en situation de mieux appréhender ces comportements, pour mieux les condamner. Il permettra enfin d'envoyer un signal clair à celles et ceux qui cherchent à contraindre une personne à renier son identité.

une union économique, mais aussi une union de valeurs. Ainsi, ce texte s'inscrit dans le combat mené depuis le début du quinquennat contre toutes les formes de discriminations et pour l'égalité des personnes LGBT+. Madame la rapporteure,

à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, madame la ministre,

de décembre, nous votions très majoritairement la création d'un délit afin d'interdire les thérapies de conversion. Celles-ci visent, dans les faits, à imposer l'hétérosexualité aux personnes LGBT. Madame la ministre, vous l'avez rappelé, être soi ne peut pas être un crime. Non, l'homosexualité ou la transidentité ne sont pas des maladies que l'on peut soigner, et non, il n'y a rien à guérir. La navette parlementaire arrive à son terme, et ce sera une nouvelle fois « oui » pour mon groupe, afin de mettre fin à ces pratiques diverses qui portent toutes atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine. Qu'elles soient biologiques, psychologiques ou confessionnelles, qu'elles soient réalisées par hypnose, hormones, électrochocs, séances d'exorcisme ou mariage forcé, celles-ci seront désormais constitutives d'un délit bien défini et spécifique,

Il existe actuellement des moyens juridiques indirects pour réprimer ces thérapies : le harcèlement, la discrimination, le viol, la torture. Il existera désormais un délit spécifique dans le code pénal, qui nommera exactement ce que subissent les victimes, ce qui est important, et permettra une plus grande célérité, grâce à une qualification directe du fait. Ce texte va dans le sens de ce que préconisait le Parlement européen en 2018, comme Mme de La Gontrie l'a rappelé à l'instant. Mon groupe votera donc les conclusions de cette commission mixte paritaire. Une fois le texte promulgué, le fait de chercher à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et d'altérer ainsi sa santé physique ou mentale, sera poursuivi en tant que tel. sera poursuivi en tant que tel. Sont exclus de ce champ les propos qui invitent simplement à la prudence, à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. L'objectif du législateur n'est évidemment pas de priver les personnes de l'accompagnement qu'elles sollicitent. Notre rapporteure a souhaité le rappeler par cette précision. Je salue d'ailleurs son travail. Elle a compris dès la première lecture l'esprit et la nécessité de ce texte.

Parler de thérapies de conversion en France en 2021 peut sembler surprenant tant ces pratiques moyenâgeuses sont barbares et contraires à nos valeurs et à nos droits fondamentaux.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les thérapies de conversion, expression générique née aux États-Unis en 1950, sont des pratiques de natures diverses, qui se fondent toutes sur des croyances selon laquelle l'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne peuvent et doivent, le cas échéant, être changées. Ces pratiques prétendent transformer une personne gay, lesbienne, bisexuelle en une personne hétérosexuelle ; transformer une personne trans ou de genre variant en une personne cisgenre. La nature dégradante des thérapies de conversion crée un environnement déshumanisant pour les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente. Il s'agit notamment de pressions psychologiques, familiales ou non, religieuses ou non, de violences physiques, de l'obligation de consulter un psychologue, d'injections d'hormones, de prescriptions d'anxiolytiques, de retraites spirituelles. Autrement dit, une personne, par des pressions, se verra contrainte de se rendre chez un psychologue pour s'entendre dire : « Vous n'êtes pas qui vous prétendez être. » Il s'agit là d'une impardonnable atteinte à l'intime liberté d'une personne. Ce principe de liberté, si cher à notre démocratie, nous devons l'affirmer pleinement pour toutes les personnes victimes des thérapies de conversion. Cette proposition de loi loi vient poser un interdit clair, même s'il est vrai que des outils juridiques existent déjà, puisque les thérapies de conversion pouvaient être réprimées par plusieurs infractions avec la circonstance aggravante aggravante d'être commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime : violences volontaires, délit d'abus de faiblesse, harcèlement moral, ou encore exercice illégal de la médecine. La création d'une infraction spécifique au sein du code pénal envoie un signal fort aux victimes puisque la loi devient plus lisible, ce qui permettra de favoriser les dépôts de plainte afin de réparer les souffrances physiques et psychologiques qu'elles ont subies. de loi, la France rejoint plusieurs pays européens ayant déjà légiféré sur le sujet, comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Si la reconnaissance de la souffrance et des conséquences particulièrement désastreuses que peuvent avoir les thérapies de conversion sur les individus est essentielle, nous devons rester vigilants concernant les mineurs qui pourraient être concernés par ce texte. Je souligne la modification apportée par le Sénat, qui a précisé que cette nouvelle infraction n'est pas constituée quand les propos ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne

faire preuve en la matière de beaucoup de prudence, notamment envers les jeunes. Nombre de psychologues, de praticiens médicaux, et notamment ceux qui sont au contact des plus jeunes, nous demandent, à nous législateurs, de ne pas copier ce qui s'est fait dans un certain nombre de pays, comme le Canada, où la loi a permis à des adolescents en recherche d'identité, souvent en grande souffrance, de changer de sexe. Car souvent, en grandissant, ceux-ci le regrettent et souhaitent faire machine arrière. Madame la ministre, mes chers collègues, nous devons résister à la montée en puissance d'un certain nombre d'associations militantes, organisées, très actives sur les réseaux sociaux, souvent agressives, quelquefois menaçantes, qui, au nom d'une forme de liberté absolue et débridée, risquent de déconstruire ce qui fait le vivre-ensemble d'une société, c'est-à-dire le dialogue, un cadre et des repères. Les élus du groupe Les Indépendants - République et Territoires voteront

Ainsi, en plus de marquer un interdit clair s'agissant des pseudo-thérapies que sont les thérapies de conversion, la loi opère une nette distinction entre thérapies de conversion et simples propos invitant à la prudence ou à la réflexion. Cette précision est bienvenue, car tout propos ne peut ni ne doit tomber sous le coup de la loi pénale. Les dispositions interprétatives ainsi introduites par la commission aux articles 1 et 3 devront permettre à la justice de faire la part des choses entre ce qui relève de l'infraction pénale et ce qui constitue des conseils ou une simple invitation à la prudence. Nous saluons également les clarifications effectuées à l'article 2 sur l'initiative du Sénat et conservées en CMP. La suppression des dispositions assimilant les infractions commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre aux infractions commises en raison de celles-ci conduira en toute logique le juge à faire application de l'infraction autonome pour punir ces faits très spécifiques. Conformément au droit positif, le procureur de la République sera toujours libre d'engager des poursuites pour plusieurs motifs dans l'hypothèse où le mis en cause aurait commis plusieurs infractions.

je me réjouis naturellement qu'un accord ait été trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur un texte d'une portée à la fois réelle, mais aussi symbolique, majeure, pour interdire ce que d'aucuns appellent des « thérapies de conversion » dans notre pays.

ce sont des tortures. Elles existent, certes, du fait d'un droit mal adapté, mais aussi et, surtout, de notre modèle de société et des violences à l'encontre des minorités

un message au parlement polonais. La semaine dernière, la Diète, chambre basse polonaise, a adopté un projet de loi visant à « protéger les enfants de la corruption morale En réalité, il s'agit d'un nouveau texte pour restreindre encore le travail des différentes associations dans les écoles, notamment des ONG qui, à rebours de l'agenda réactionnaire et LGBTphobe du gouvernement, vont à la rencontre des élèves, font leur éducation sexuelle, leur parlent de la diversité et les éduquent à la tolérance et à l'acceptation de soi.

qu'elles et ils ne sont pas seuls, qu'elles et ils ont toute leur place dans ce monde, dans cette Europe, comme elles et ils sont. Je veux leur dire qu'il y a partout en Europe des personnes, mais aussi des élus, des parlements qui sont de leur côté et qui le seront toujours. C'est dans cet esprit que le groupe écologiste votera évidemment ce texte. Nous appelons plus généralement à un sursaut européen pour la protection de l'État de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales, dont la violation touche en premier lieu les minorités, en particulier les personnes LGBTI. La parole

En 2015, un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme appelait à l'interdiction des thérapies de conversion, qualifiées à juste titre de « pratiques contraires à l'éthique, dénuées de fondement scientifique, inefficaces et, pour certaines d'entre elles, constitutives de torture ».

l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sera condamné. Et nous sommes satisfaits, malgré des attaques en première lecture, que l'identité de genre soit bel et bien intégrée et que la transidentité, même des mineurs, soit reconnue et protégée. La création d'un délit spécifique est, pour nous, nécessaire pour mieux combattre ces pratiques inhumaines et mieux quantifier les victimes. Celles-ci présentent de grandes souffrances. Certaines ont subi de véritables tortures, souvent mal identifiées et peu sanctionnées. Les travaux du Sénat n'ont pas dénaturé le texte de l'Assemblée nationale, en conservant notamment l'extension des cas d'aggravation des peines et la possibilité pour les associations de se porter partie civile en cas d'agression homophobe, lesbophobe ou transphobe. Aussi notre assemblée a-t-elle adopté le 7 décembre dernier à une large majorité cette proposition de loi en lui apportant plusieurs améliorations, également conservées par la commission mixte paritaire. Je pense notamment à l'obligation, à l'article 1, pour le juge pénal, en cas de condamnation d'un parent, de s'interroger sur le retrait ou non de l'autorité parentale et à l'ajout, à l'article 3, d'une circonstance aggravante si la victime est mineure ou s'il s'agit d'une personne vulnérable. Finalement, ce texte de consensus honore nos deux chambres et enverra un signal fort, en marquant le refus par la représentation nationale des pratiques d'un autre âge et la nécessité de protéger celles celles et ceux qui en seraient encore victimes. Cependant, mes chers collègues, tout en approuvant sans réserve ce nouveau dispositif de sanction, qui vient inscrire dans notre droit un interdit plus que nécessaire, nous nous devons de souligner que la protection de ces personnes ne sera effective que si ce mécanisme de répression est combiné à une mesure forte de prévention et de lutte contre les violences dont sont victimes les personnes LGBTQIA+. Une telle mesure n'est pas tout à fait au point et nécessite, contrairement au dispositif punitif mis en place, des moyens. Or c'est toujours cette question qui fait la différence entre les paroles et les actes. Au demeurant, le chemin, bien qu'entamé, est encore long vers l'éradication de toute forme de discriminations pouvant aller jusqu'à ce genre de pratiques. C'est pourquoi tous les moyens doivent être engagés dans la lutte contre les discriminations de nos concitoyennes et concitoyens LGBTQIA+. Pourquoi d'ailleurs ne pas en faire l'une des grandes causes nationales du prochain quinquennat ? Je lance l'idée à toutes les candidates et à tous les candidats à quelques mois de l'élection présidentielle. Il est important à cet égard d'écouter les associations travaillant sur de tels sujets, d'entendre leur parole

dans une société où chacune et chacun, dans sa diversité, peut pleinement s'épanouir. La République et ses valeurs gagneront à respecter cette société multiple. Pour toutes ces raisons, nous voterons les conclusions de la CMP sur la présente proposition de loi. La parole

la proposition de loi, dont l'examen touche aujourd'hui à sa fin, vise à poser un interdit clair concernant des pratiques qui prennent des formes variées, mais qui ont toujours des conséquences dramatiques sur la santé et sur le bien-être des personnes qui y sont soumises. Ces pratiques sont souvent désignées, par commodité, par l'expression « thérapies de conversion », bien que l'orientation sexuelle et la transidentité ne soient en aucun cas- cela a été souligné -des maladies. Si c'est désormais un acquis de notre société et si nous sommes heureusement loin du postulat archaïque selon lequel l'homosexualité et la transsexualité seraient des déviances à corriger, il faut que cela soit inscrit dans la loi : il n'y a rien à guérir. On relate de véritables actes de torture, particulièrement cruels, qui doivent être condamnés, pénalement condamnés. Qu'elles s'inscrivent dans un contexte pseudo-médical ou au sein d'un mouvement religieux, qu'il s'agisse de médicaments, d'électrochocs ou même de séances d'exorcisme, toutes ces pratiques suscitent une profonde souffrance chez ceux qui les subissent. Dès lors que le débat sur l'homosexualité et le genre cesse d'être tabou, le voile se lève également sur des pratiques d'un autre âge ayant conduit tant de jeunes au désespoir, et même au suicide. Nous saluons donc la présente proposition de loi, qui permettra de clarifier définitivement l'interdiction des thérapies de conversion. Les travaux sur ce texte sont un bon exemple de travail parlementaire apaisé et efficace. Le Sénat a préservé les apports de l'Assemblée nationale, qui a respecté ceux du Sénat. Ce consensus honore nos deux chambres et permettra de protéger au plus vite les personnes visées par ces fameuses thérapies de conversion. Remercions encore notre collègue députée Laurence Vanceunebrock d'avoir déposé ce texte tant attendu, qui permettra d'empêcher qu'il y ait de nouvelles victimes. Les débats au Sénat ont surtout porté sur la prise en compte de l'identité de genre, certains collègues craignant que l'adoption du texte n'empêche des parents ou des professionnels de santé de recommander une attitude de prudence, particulièrement face aux demandes d'adolescents souhaitant s'engager dans un parcours de transition. Il est clair qu'une telle décision doit être mûrement réfléchie et qu'elle ne peut pas être prise sous le coup d'une impulsion, les tumultes de l'adolescence ne permettant pas toujours d'éclairer les décisions. Dans l'intérêt prioritaire des personnes décidant de changer de sexe, il faut impérativement veiller à ce que de telles décisions sans retour ne soient jamais regrettées. Sinon, là encore, que de souffrances, que de douleurs Pour apaiser ces craintes et sécuriser la phase de conseil, le Sénat a ajouté aux articles 1 et 3 des dispositions interprétatives pour préciser qu'une simple invitation à la prudence et à la réflexion adressée à une personne envisageant de s'engager dans un parcours de transition ne saurait constituer une infraction. Le groupe Union Centriste se félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord le 14 décembre dernier. Je remercie tout particulièrement notre collègue Dominique Vérien du travail réalisé, à la fois précis et empathique, Nous soutiendrons ce texte équilibré et respectueux des apports du Sénat. Je termine mon propos en formulant le souhait que le respect des identités de genre et des orientations sexuelles, désormais gravé dans le marbre en droit français, dépasse le cadre de nos frontières nationales que nulle part dans le monde, aucun parent, aucun thérapeute, aucun gouvernement, aucune religion n'ait le droit de donner ou de faire donner par la force ce qu'une victime a appelé des « leçons d'amour » ! La parole

Notre droit devrait donc bientôt permettre de sanctionner les thérapies de conversion. Ces pratiques, si elles pouvaient être sanctionnées au motif de l'abus de faiblesse, ne permettaient pas une reconnaissance complète des victimes. Aussi, nous nous réjouissons de l'instauration future d'un délit spécifique interdisant les thérapies de conversion et les punissant de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Au-delà, ce texte vient poser un véritable interdit social et permettra de faciliter la prise en charge des victimes. C'est un souhait qu'avait exprimé le groupe du RDSE depuis longtemps. Comme l'avait rappelé mon collègue Jean-Yves Roux lors de l'examen du texte, nous sommes depuis longtemps mobilisés sur cette question. 2019, notre ancienne collègue Françoise Laborde avait déposé une proposition de loi visant à engager une campagne de prévention et de lutte contre les thérapies de conversion. Voilà quelques mois encore, par l'intermédiaire de Christian Bilhac, nous déposions un amendement- il a, hélas ! été déclaré irrecevable -lors de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République ; il visait à créer une infraction autonome réprimant les thérapies de conversion. Vous comprendrez donc notre satisfaction. Certes, sur un tel sujet, les risques étaient grands, au regard non pas du texte que nous avions adopté en commission, puis en séance, mais de ce qu'avaient souhaité certains collègues des amendements visant à supprimer du champ du dispositif l'identité de genre d'une personne. Nous n'avions pas fait l'erreur d'adopter une position restreignant le champ de la nouvelle infraction que crée ce texte. Je m'en réjouis, car le champ de l'infraction proposée ne doit pas être restreint, sachant surtout combien ces pseudo-thérapies peuvent prendre des formes multiples thérapies non scientifiques, stages, conférences, entretiens, qui peuvent être accompagnés d'injections de testostérone, de traitements par électrochocs ou encore de diffusions d'images et de vidéos afin de formater les esprits.

À ce titre, la série d'entretiens proposés par un grand hebdomadaire national ces derniers jours est édifiante. Elle revient sur la lente et difficile acceptation de l'homosexualité dans notre pays, sur la vie clandestine d'avant 1982, avec ce qu'on appelait les « paniers à salade », où des homosexuels étaient placés en garde à vue d'autres étaient même détenus pour « outrage public à la pudeur commis sur personne de même sexe ». Oui, cette histoire est ancienne, mais quarante après l'abrogation du délit d'homosexualité, des discriminations perdurent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, on ne peut qu'accueillir avec satisfaction le texte établi par la commission mixte paritaire. Les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont désormais clairement identifiées comme des délits. Cette proposition de loi permettra de mieux protéger les victimes de ces actes barbares et, je l'espère, de libérer la parole sur un phénomène peu publicisé, pourtant à l'origine de souffrances terribles. Certes, une telle avancée est donc positive. Mais Mais le fait que ces thérapies subsistent encore en 2022 est révélateur des problèmes sous-jacents que doivent encore affronter toutes les personnes qui s'émancipent du cadre binaire et hétéronormé dominant notre société. Vivre une sexualité libre et choisir son identité de genre sont des droits absolus. Il est important de le dire et de le répéter. Pourtant, ces droits sont aujourd'hui menacés. Au sein de notre communauté européenne, certains pays s'acharnent à mettre en place en place des politiques excluantes et stigmatisantes à l'encontre des personnes LGBTQIA+. En France, la menace à l'encontre de cette population est de plus en plus pesante. J'en veux pour preuve les résultats d'un sondage

Moins de 20 % des victimes décident de porter plainte. Les propos tenus à l'encontre de la communauté LGBTQIA+ par un candidat à l'élection présidentielle dont je tairai le nom au sein de cette honorable assemblée ne font qu'exacerber ce climat de violence et d'insécurité. Face à de tels dangers, nous ne pouvons pas nous contenter des acquis de la proposition de loi. Nous devons continuer notre travail de lutte contre l'homophobie et les discriminations liées au genre. Il faut accroître les interventions en milieu scolaire pour prévenir et et éduquer. La formation des professionnels de santé, de police et de justice doit être développée. Soutenir les victimes de violences homophobes et de discriminations à la fois psychologique et juridique devrait être une priorité. Je voterai donc pour ce texte et je vous assure de ma détermination à poursuivre le travail nécessaire à la protection et au développement des droits des personnes LGBTQIA+.

En France, comme dans le monde entier, ce terme a été popularisé et forgé par quelques figures médiatisées. Le nom d'Irène Frachon évoque immédiatement l'affaire du Médiator, celui d'Edward Snowden, les écoutes de la NSA, et, plus récemment, Frances Haugen, le traitement des informations par certains réseaux sociaux. Ces femmes et ces hommes se sont distingués, parce qu'ils ont découvert avant d'autres un risque. Ils ont dénoncé des pratiques qu'ils estimaient illicites ou ils ont révélé des faits qui méritaient d'être portés dans le débat public. Ils ont agi par devoir, en conscience, ou pour défendre l'intérêt général. Mais ils ont aussi heurté des intérêts particuliers, parfois puissants. Leurs révélations ont pu mettre en cause les organisations dans lesquelles ils travaillaient ou avec lesquelles ils sont en contact ; pour cela, elles les exposent à des risques de représailles. Discriminés, licenciés, parfois poursuivis en justice, certains d'entre eux vivent alors des mois, voire des années de difficultés professionnelles et, parfois, de drames personnels. De telles situations ne sont pas le sort des seules figures médiatisées. Régulièrement, des salariés, des fonctionnaires ou des citoyens sont témoins d'infractions ou de menaces sur l'intérêt général et sont confrontés à un dilemme bien connu : se taire et laisser prospérer, ou parler et risquer des représailles. C'est ce dilemme que la protection des lanceurs d'alerte vise à surmonter. Cette protection est l'enjeu du projet de loi et du projet de loi organique qui sont aujourd'hui en discussion devant vous après avoir devant vous après avoir été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Sans permettre une protection effective, sans organiser des garanties réelles et efficaces, un texte sur les lanceurs d'alerte ne serait rien d'autre qu'un dispositif procédural creux

aux lanceurs d'alerte. Le défi de la protection des lanceurs d'alerte est immense et complexe. La révélation de dangers ou de faits délictueux se fait le plus souvent au bénéfice du bien commun, mais certaines dénonciations peuvent également se révéler malhonnêtes ou malveillantes. La frontière entre le lanceur d'alerte et le délateur doit donc être impérativement et très clairement tracée. Mal calibrées, vagues ou trop ouvertes, les conditions donnant droit à une protection légitime pourraient contribuer à faire émerger une société de la suspicion, du tous contre tous. Sur ce point également, le Gouvernement s'exprimera tout à l'heure pour que des conditions et une définition claires permettent de tracer une frontière juste et dénuée d'ambiguïté. Un texte sur les lanceurs d'alerte est ainsi le lieu d'un équilibre délicat : il s'agit d'organiser un cadre pour recueillir efficacement les alertes, sans encourager les règlements de comptes ; d'accorder une protection effective, mais seulement pour les comportements vertueux. Le travail législatif entrepris dans le cadre de ces deux propositions de loi constitue la transposition d'une directive européenne, mais les textes que nous allons examiner ne partent pas d'une feuille blanche. La France a été pionnière. Elle s'est d'abord progressivement dotée de nombreux dispositifs spécifiques permettant de lancer des alertes sur des sujets particuliers, par exemple en matière financière ou de harcèlement au travail.

C'est ce texte qui sert de socle aux améliorations prévues par les propositions de loi que nous allons examiner. Enfin, l'Union européenne a adopté la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Grâce au soutien actif

européennes. Dans ce contexte, le député Sylvain Waserman a déposé deux propositions, l'une organique et l'autre ordinaire, et l'Assemblée nationale a adopté un texte ambitieux et équilibré, construit en lien avec l'ensemble des parties prenantes, tout en conservant le souci d'une juste transposition des dispositions de la directive. C'est dans cette recherche de l'amélioration du texte que se sont inscrits vos travaux. Madame la rapporteure, nous avons suivi à quel point vous vous êtes engagée au sein de la commission des lois sur ce texte. Votre action a permis d'améliorer un certain nombre de rédactions, dans le respect du cadre européen. Même si certains aspects du texte devraient encore pouvoir être ajustés, comme nous le verrons au cours de son examen, ces améliorations et l'état d'esprit constructif dans lequel nous travaillons ensemble permettront, j'en suis sûre, d'aboutir à l'adoption d'un texte clair et équilibré. J'aborderai à présent quelques aspects marquants de ces textes et des avancées importantes qu'ils permettent d'abord d'inscrire dans notre droit les avancées de la directive européenne. Certaines d'entre elles méritent une attention particulière. Une première évolution porte sur l'accessibilité des procédures d'alerte. Actuellement, le droit français est fondé sur l'idée qu'une alerte est toujours traitée plus efficacement en interne par l'organisme directement concerné. Cette idée n'est pas dépourvue de fondement, mais elle a sans doute été inscrite de manière excessive dans le droit français. Celui-ci fait fait obligation à un lanceur d'alerte de s'adresser d'abord à son employeur. Ce n'est qu'en l'absence de diligences de ce dernier ou en cas de danger grave et imminent que le lanceur d'alerte peut porter son alerte devant l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou un ordre professionnel. telle hiérarchie entre l'alerte interne et externe soulève deux difficultés majeures. D'abord, obliger en principe le lanceur d'alerte à s'adresser à son supérieur peut l'exposer à un risque accru de représailles, surtout dans les petites structures. Ensuite, les critères prévus pour faire usage du canal externe sont complexes et peu connus en pratique. Cette complexité a pu priver certains lanceurs d'alerte de bonne foi de la protection qu'ils auraient pourtant méritée. La directive, reprise à l'article 3 de la proposition de loi ordinaire, permet d'abandonner une telle hiérarchie des canaux et assure donc une protection plus complète des lanceurs d'alerte. Mais elle n'abandonne pas pour autant l'idée qu'une alerte est mieux traitée en interne. interne. Elle demande en effet d'encourager le recours à un canal interne lorsque celui-ci est plus efficace, ce qui sera fait au niveau réglementaire, notamment en assurant une publicité active de ce canal auprès des salariés et des agents. Une deuxième avancée européenne procède de l'extension de la protection au-delà du seul lanceur d'alerte : désormais, ses proches, ses collègues, les personnes morales qui lui sont liées et quiconque l'aide au cours de la procédure- en d'autres termes, les « facilitateurs » de l'alerte -pourront bénéficier de la même protection. Cette extension permet d'offrir un véritable cercle de protection au lanceur d'alerte et de rompre son isolement. Les propositions de loi soumises à votre examen, mesdames, messieurs les sénateurs, ne se limitent pas à la seule transposition de cette directive. Pour le Gouvernement, elles doivent aussi permettre d'inscrire dans notre droit des avancées supplémentaires, ambitieuses et significatives, répondant aux attentes exprimées par la société civile.

externes. Nous serons donc favorables au rétablissement d'une définition unique permettant d'accéder à la protection du lanceur d'alerte. En outre, les autorités externes seront clairement identifiées par décret en Conseil d'État, de façon à ce que le lanceur d'alerte sache à qui s'adresser.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la directive européenne nous a placés devant l'obligation d'améliorer sur quelques points précis, et dans un champ restreint, notre dispositif général d'alerte. Les présentes propositions de lois organique et ordinaire nous offrent l'occasion d'aller au-delà de ces quelques exigences,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les lanceurs d'alerte sont des personnes qui, dans l'intérêt de la société, révèlent des informations portant sur des crimes, des délits, et plus généralement sur des violations de règles de droit ou sur d'autres faits allant à l'encontre de l'intérêt général. Les lanceurs d'alerte jouent un rôle essentiel dans notre démocratie, pour mettre au jour des scandales, faire réprimer des infractions et faire progresser le débat public. Sans le courage d'Irène Frachon, pour ne prendre qu'un exemple, le scandale du Mediator n'aurait pas eu lieu. Nous avons donc le devoir de protéger les lanceurs d'alerte contre les conséquences éventuelles de leurs actes. Car, en révélant des informations sensibles, les lanceurs d'alerte peuvent s'exposer à des mesures de représailles. Ils peuvent également voir leur responsabilité engagée, pour avoir porté atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité, ou en raison des dommages qu'ils peuvent avoir causés. La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a eu le mérite de créer un régime général de protection des lanceurs d'alerte. Mais celui-ci doit encore être amélioré. La transposition de la directive du 23 octobre 2019 nous en donne l'occasion. La commission des lois a examiné le 15 décembre dernier les propositions de loi organique et ordinaire dont nous sommes saisis aujourd'hui, deux textes dont l'initiative revient à notre collègue député Sylvain Waserman, que je salue. La commission les a accueillis favorablement, tout en y apportant un certain nombre de modifications. Depuis le mois de décembre, nous avons été soumis à un intense lobbying de la part d'associations, les unes très respectables, les autres beaucoup moins, qui nous ont accusés d'avoir « détricoté » les deux textes, et même d'avoir imposé un retour en arrière par rapport à la loi Sapin II. Ces accusations sont, pour l'essentiel, sans fondement, et elles reposent sur une lecture hâtive des textes issus de la commission. Il me paraît donc nécessaire de procéder à quelques mises au point. La protection des lanceurs d'alerte doit reposer sur un équilibre. le législateur doit protéger ceux qui lancent l'alerte à bon escient, il ne peut pas faire abstraction des autres intérêts légitimes qui sont en cause. Nous devons veiller, notamment, à ce que les secrets protégés par la loi ne soient pas trop facilement éventés et à ce que la réputation des personnes physiques et morales ne soit pas ternie par des alertes abusives ou infondées. En adoptant la loi Sapin II, le législateur français avait recherché ce juste équilibre. Mais cette loi, je l'ai dit, doit être améliorée, car elle souffre de trois défauts principaux, mis en évidence dans un rapport transpartisan des députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix. En premier lieu, la loi exige que le lanceur d'alerte agisse de manière « désintéressée », ce qui est trop vague et laisse une marge d'appréciation excessive au juge. La proposition de loi supprime donc ce critère de désintéressement, ce que la commission des lois a approuvé. En deuxième lieu, le régime actuel impose en principe au lanceur d'alerte d'effectuer d'abord un signalement en interne, au sein de son organisation, avant de s'adresser à une autorité externe. En dernier ressort, il est autorisé à divulguer publiquement les faits. La hiérarchisation des canaux de signalement interne et externe pose problème, d'abord parce que beaucoup d'entreprises et d'administrations n'ont pas mis en place la procédure de recueil des signalements prévue par la loi, ensuite parce que le lanceur d'alerte peut s'exposer en interne à des mesures de représailles. Conformément à la directive, les députés ont prévu que les lanceurs d'alerte puissent désormais s'adresser directement à une autorité externe, sans passer par le canal interne. C'est un choix judicieux, auquel la commission des lois a souscrit. En troisième lieu, la loi Sapin II ne prévoit pas de mesures d'accompagnement juridique et financier suffisantes au bénéfice des lanceurs d'alerte. L'Assemblée nationale a essayé de combler cette lacune, malgré les contraintes de l'article 40 de la Constitution. Nous avons approuvé la plupart des mesures proposées, sauf lorsqu'elles se heurtaient à des obstacles juridiques insurmontables. Si l'Assemblée nationale s'était contentée d'apporter ces correctifs nécessaires à la loi Sapin II, nous n'aurions rien eu à y redire. Mais ce n'est pas exactement ce qu'ont fait les députés Leur tâche était difficile, puisqu'ils devaient à la fois procéder aux améliorations de la loi Sapin II préconisées par le rapport Gauvain-Marleix et transposer exhaustivement la directive de 2019. Or cette directive définit un régime de l'alerte assez sensiblement différent du régime actuel de droit français sur des points importants, alors même que son champ matériel d'application est beaucoup plus limité, puisqu'elle ne concerne que la violation de certaines règles de droit européen. C'est également un texte touffu, mal rédigé, et qui comprend bon nombre d'ambiguïtés. Pour l'essentiel, les députés ont fait le choix d'appliquer les solutions de la directive à l'ensemble des informations qui relèvent aujourd'hui du régime de l'alerte en droit français. Même dans le champ d'application spécifique à la directive, ils ont été au-delà de ce que celle-ci exige. Sur certains points, les choix de l'Assemblée nationale nous ont paru devoir être réexaminés. Nous y reviendrons en détail au cours de l'examen des articles, mais je veux dès à présent insister sur trois éléments. Premier point : la nature des informations susceptibles d'être signalées ou divulguées dans le cadre d'une alerte. La loi Sapin II protège les personnes qui révèlent des faits graves : un crime, un délit, toute autre violation grave d'une règle de droit, ou encore une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général. Le législateur français, en 2016, avait estimé que seule la révélation de faits suffisamment graves pouvait justifier de porter atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité. Or la directive, dans son champ d'application bien défini, supprime ce critère de gravité. Compte tenu du fait que la loi française a un champ d'application beaucoup plus vaste, et même indéfini, la commission des lois a estimé nécessaire de maintenir ce critère de gravité, sauf dans le champ de la directive. Nous avons suivi en cela l'avis du Conseil d'État. Sur ce sujet précis, il ne nous a paru ni nécessaire ni opportun de surtransposer la directive. Deuxième point : les conditions dans lesquelles un lanceur d'alerte peut divulguer publiquement les informations dont il dispose, par exemple par voie de presse ou sur les réseaux sociaux. C'est un sujet particulièrement important, puisque c'est au moment de la divulgation publique des informations que l'atteinte aux secrets protégés et à la réputation des personnes mises en cause est la plus forte. Il est normal qu'un lanceur d'alerte puisse révéler les faits au public s'il a d'abord effectué un signalement auprès de l'autorité compétente sans obtenir de réponse satisfaisante. Il est également normal qu'il puisse le faire si la saisine de l'autorité externe l'expose à des risques de représailles ou ne présente aucune chance de succès, par exemple en raison d'une collusion entre l'autorité externe et l'auteur des faits. Enfin, et c'est le troisième cas, il est parfaitement légitime que le lanceur d'alerte puisse divulguer les informations dont il dispose, sans attendre la réponse d'une autorité, lorsqu'il existe un danger grave et imminent, ou en présence d'un risque de dommages irréversibles. C'est ce que prévoit la loi Sapin II. Mais la directive supprime, dans ce troisième cas, le critère lié à la gravité du danger, et elle autorise la divulgation publique d'informations sans signalement préalable en cas de danger soit soit imminent, soit manifeste. À vrai dire, le texte de la directive sur ce point est à peu près incompréhensible ... Soyons clairs : pour la commission, seul un danger imminent, manifeste et d'une gravité suffisante justifie de court-circuiter la procédure normale de signalement à l'autorité compétente. Nous avons beau vivre au temps des hashtags #BalanceTonMaire ou #BalanceTonPatron, il existe en France des autorités administratives et judiciaires qui ont pour mission de prendre en charge les signalements, de mener des enquêtes et d'imposer des sanctions ou d'autres mesures correctrices, sans qu'il soit nécessaire de déballer systématiquement sur les réseaux sociaux ou dans la presse n'importe quelles informations. Troisième point : la protection des facilitateurs, c'est-à-dire des personnes qui aident les lanceurs d'alerte dans leurs démarches. À ce sujet, le débat est devenu extrêmement confus. Les personnes qui assistent les lanceurs d'alerte sont déjà indirectement protégées par les dispositions qui protègent les lanceurs d'alerte eux-mêmes, notamment en matière pénale. Le principal intérêt du nouveau statut de facilitateur, c'est d'étendre aux personnes concernées l'interdiction de certaines mesures de représailles. Or, pour la plupart d'entre elles, les mesures de représailles interdites ne peuvent viser que des personnes physiques. C'est la raison pour laquelle la directive ne prévoit d'accorder le statut de facilitateur L'Assemblée nationale a fait le choix d'y ajouter les personnes morales à but non lucratif. Ce choix a suscité beaucoup d'inquiétudes, plus ou moins fondées, et c'est pourquoi la commission, à titre conservatoire, a fait le choix de revenir sur ce point à une stricte transposition de la directive. Je ne pense pas que nos divergences avec les députés soient insurmontables et j'ai bon espoir que nous parvenions à un accord en commission mixte paritaire. Je veux néanmoins insister, pour finir, sur un point de vigilance, qui concerne l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte et des facilitateurs. Aujourd'hui, en droit français, les lanceurs d'alerte ne peuvent être poursuivis pénalement pour avoir porté atteinte à un secret protégé par la loi s'ils ont respecté les conditions de fond et de procédure prévues pour bénéficier du régime de protection. Le texte de l'Assemblée nationale prévoit d'étendre cette irresponsabilité pénale à des infractions connexes, puisqu'il vise également le fait d'avoir « soustrait » des données couvertes par le secret ou des données confidentielles. La portée exacte de cet ajout est assez incertaine. On ne sait pas bien à quelles infractions connexes l'irresponsabilité s'étendrait : vol de documents, abus de confiance ? En signe de bonne volonté, la commission n'a pas voulu supprimer cet ajout, mais elle a estimé indispensable d'apporter des précisions pour dissiper les inquiétudes très vives que le texte de l'Assemblée nationale a suscitées, notamment dans le monde agricole. Je veux rappeler le contexte. Une certaine association animaliste, qui se prévaut indûment de la qualité de lanceuse d'alerte, vient d'être condamnée pénalement pour violation de domicile. Ses militants n'hésitent pas à s'introduire dans des élevages à l'insu des propriétaires, à y prendre des images, puis à les diffuser, de manière plus ou moins tronquée, sur les réseaux sociaux. Ces agissements sont proprement inadmissibles. S'autoproclamer défenseur de l'intérêt général n'autorise pas tout. La commission a donc tenu à inscrire expressément dans la loi que l'irresponsabilité pénale prévue au bénéfice des lanceurs d'alerte et des facilitateurs ne s'étend pas aux atteintes à la vie privée la vie privée et aux systèmes de traitement automatisé de données, qui font l'objet d'incriminations spécifiques dans le code pénal. Nous verrons s'il est possible de parvenir à une rédaction plus simple, mais nous ne transigerons pas sur l'objectif. Protéger les lanceurs d'alerte, ce n'est pas laisser place à la loi de la jungle ni autoriser de prétendus justiciers à avoir recours à des méthodes de délinquants. La parole est à Mme

à l'heure où des citoyens en mal de reconnaissance s'autoproclament lanceurs d'alerte du fin fond de leur canapé, il nous paraît bien utile de revenir à une définition juridique harmonisée à l'échelle européenne et à l'État de droit. Lanceur d'alerte n'est assurément pas un titre de gloire personnelle : il s'agit d'un combat étayé, exigeant, solitaire, dangereux, au service de la vérité. Le statut du lanceur d'alerte était jusqu'à présent régi par les dispositions novatrices de la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II. Or l'association Transparency soulignait dès 2020, dans son rapport d'évaluation des articles relatifs aux lanceurs d'alerte, que « leur protection se heurte encore à de nombreux obstacles et [que] le parcours d'un lanceur d'alerte reste trop souvent périlleux et coûteux Elle en appelait à la transposition rapide de la directive européenne du 23 octobre 2019, qui est beaucoup plus protectrice pour les lanceurs d'alerte européens. Chers collègues, la proposition de loi Waserman de transposition de cette directive et son corollaire, la proposition de loi organique renforçant le rôle du Défenseur des droits, que nous examinons ce soir, constituent effectivement des avancées notables. Je ne reviens pas sur le détail de leurs dispositions. Au mois de décembre dernier, notre commission a proposé quelques avancées auxquelles nous souscrivons, notamment l'extension du bénéfice de la protection aux facilitateurs, ainsi que la création d'un adjoint au Défenseur des droits. Pourtant, d'autres propositions nous paraissent en retrait par rapport à la proposition de loi initiale, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Nous avons ainsi déposé un amendement afin de revenir à la définition initiale du lanceur d'alerte,

Nous souhaitons de la même manière réintroduire la possibilité pour des personnes morales à but non lucratif d'avoir la qualité de facilitateur. Mes chers collègues, le lanceur d'alerte est seul, profondément seul. Se priver de l'appui de syndicats ou d'associations, c'est le plus sûr moyen pour lui de voir son action ne pas aller au bout. Enfin, nous avons souhaité réintroduire la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent ou manifeste. Le temps de saisine et d'examen du Défenseur des droits est long, jusqu'à six mois, ce qui permet d'apprécier tous les ressorts de l'alerte et d'en circonscrire les abus. Mais il peut se passer beaucoup d'événements avant la mise en oeuvre de la protection, y compris le pire. Faisons confiance à la presse, qui sait mener des enquêtes approfondies. Je terminerai par une inquiétude. La mission du Défenseur des droits est étendue, c'est une bonne chose, et je crois sincèrement que l'institution mériterait des effectifs supplémentaires. Pourtant, que peut faire le Défenseur des droits face à des campagnes de déstabilisation de lanceurs d'alerte venant de territoires extra-européens ou menées sur des réseaux privés virtuels (VPN) extraterritoriaux ? De quels outils d'intervention ou de sanctions disposons-nous réellement ?

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans une société dominée par des entreprises qui prônent le profit au détriment de l'intérêt général, le rôle des lanceurs d'alerte est devenu essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie. Notre devoir en tant que parlementaires est de protéger ces personnes, véritables héroïnes et héros de notre époque, contre les entraves et menaces qu'elles subissent, en leur garantissant un cadre juridique protecteur. C'est ce qu'avait entrepris la loi Sapin II de 2016, en établissant, entre autres, une définition légale du statut de lanceur d'alerte. Face à certaines lacunes de cette loi et au vote en 2019 d'une directive européenne visant à développer le statut de lanceur d'alerte, il était devenu nécessaire de légiférer sur le sujet. C'est ce qu'ont entrepris nos collègues de l'Assemblée nationale en déposant un texte particulièrement ambitieux, pouvant faire de la France une référence européenne sur le sujet. Je tiens à saluer le travail du député Sylvain Waserman, à qui revient l'initiative de la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui. Les avancées de cette dernière sont considérables. La définition des lanceurs d'alerte est étendue, le statut juridique pour l'entourage des lanceurs d'alerte plus inclusif, les mesures de protection renforcées. Vous le savez, ce texte a été adopté à l'unanimité par les députés. Malheureusement, cette ambition n'a pas été celle de la commission des lois du Sénat. Cette dernière s'est particulièrement appliquée à démanteler toutes les avancées du texte, au point de lui faire perdre une part importante de sa substance. La commission transgresse ainsi la directive européenne, qui

J'ai été assez surprise d'apprendre par la presse comment certaines et certains élus ont été influencés par des lobbyistes pour affaiblir cette proposition de loi, mus par la volonté de protéger les intérêts financiers de certaines entreprises. J'espère que nos débats leur permettront de revoir leur position. C'est dans notre intérêt commun. Il y va de la bonne santé de notre démocratie. La parole

nous sommes au beau milieu d'une campagne présidentielle et nous savons que cette période ne se prête pas à la bienveillance entre partis concurrents. L'examen du projet de loi sur le passe vaccinal nous a également rappelé que l'heure ne se prêtait pas davantage à la bienveillance entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les premières heures de la présidence française du Conseil de l'Union européenne nous ont enfin démontré que l'Europe constituait, comme toujours, un bouc émissaire idéal en période de campagne électorale. Aujourd'hui, nous choisissons d'aller à l'encontre de ces trois règles politiques, en vantant le consensus entre partis, en saluant le travail des députés et en louant le contenu d'une directive européenne ! Les deux textes que nous avons l'honneur d'étudier aujourd'hui sont plus que bienvenus, parce qu'ils étaient attendus. Notre pays a en effet l'obligation de transposer la directive européenne d'octobre 2019 portant sur les lanceurs d'alerte. Comme la plupart de nos partenaires européens, c'est avec retard que nous opérons la transcription de ce texte, la date limite étant fixée au 17 décembre 2021. Il faut toutefois saluer le gouvernement français qui, en inscrivant ces textes à l'ordre du jour aujourd'hui, permet à notre pays de démarrer sa présidence du Conseil de l'Union européenne en respectant ses engagements. Seuls

autrement ? C'est bien la conception française de la protection des lanceurs d'alerte, découlant de la loi Sapin II, qui a abouti à la directive que nous transposons aujourd'hui.

contient. Olivier Marleix a su expliquer de manière convaincante au Palais Bourbon, d'abord dans son rapport d'évaluation de la loi Sapin II, puis en soutien aux textes examinés aujourd'hui, la reconnaissance que nous devons à Irène Frachon, à Stéphanie Gibaud, à Antoine Deltour et aux autres lanceurs d'alerte, célèbres ou inconnus.

Même Mediapart a salué le progrès que représentaient les deux propositions de loi dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale. Le mieux étant l'ennemi du bien, madame la rapporteure, le groupe socialiste du Sénat a choisi de ne pas déposer d'amendements mieux-disants en commission, afin de préserver les acquis du texte et de permettre une adoption rapide de celui-ci. Il restait pourtant des possibilités d'améliorations, comme le recours au statut de salarié protégé ou la création d'un fonds de solidarité. Mais alors que tout le monde se félicitait de l'extension de la protection aux personnes morales à but non lucratif, de la reconnaissance des trois piliers de l'alerte, de la définition des lanceurs d'alerte et des facilitateurs, de la lutte contre les procédures bâillons et de la meilleure reconnaissance du rôle du Défenseur des droits en matière de protection, nous avons été déçus des orientations retenues par la commission des lois. En effet, les amendements adoptés en commission, sous l'impulsion probable de lobbys économiques ou de jusqu'au-boutistes du secret-défense, ne vont pas dans la bonne direction. Les réactions ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. Tout ce que ce pays compte comme lanceurs d'alerte- les mêmes que vous avez auditionnés pour rédiger votre rapport, madame contre les modifications apportées au texte de Sylvain Waserman. Le Sénat avait déjà fait obstacle à la loi sur le devoir de vigilance et n'avait guère été coopératif sur la loi Sapin II ... Chers collègues, à vous de montrer aujourd'hui que le Sénat peut se montrer à la hauteur des exigences de l'économie moderne en termes de protection des lanceurs d'alerte. Le XXI siècle sera sévère avec ceux qui tentent d'esquiver les nouveaux standards. Ceux-ci sont indispensables pour faire face aux exigences d'une économie dont les acteurs doivent être à la hauteur de la transition climatique et écologique, aux conséquences de l'émergence du numérique et aux risques de l'exploitation de la donnée, au respect de la dignité et des droits de chacun, partout, dans une économie globalisée. Nous avons la conviction que les entreprises qui jouent le jeu de la mise en place de dispositifs d'alerte interne sont souvent mieux protégées et plus efficaces que celles qui cherchent à esquiver leurs obligations. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, le groupe socialiste décidera de son vote en fonction du sort qui sera réservé aux amendements de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale, qui a su faire consensus. Madame la rapporteure, nous avons noté votre évolution entre l'examen du texte en commission et sa discussion en séance. Nous saluons ce mouvement, probablement dû aux alertes reçues dans l'intervalle. du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaitent que cette séance parachève cette évolution et permette d'aboutir aussi rapidement que possible à un texte consensuel.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la nécessité et l'opportunité des textes organique et ordinaire que nous examinons aujourd'hui peuvent être admises sans difficulté. premier lieu parce que la France doit transposer une directive de l'Union européenne du 23 octobre 2019, qui implique de mettre à niveau notre droit national relatif aux lanceurs d'alerte

Or chacun sait que cet objectif de transposition impose de légiférer suffisamment vite au regard des délais, déjà dépassés, dont nous disposons pour le faire. Ces propositions de loi s'imposent, ensuite, à la lumière des travaux approfondis dont elles constituent l'aboutissement.

Ils ont mis en évidence le bilan mitigé de la mise en oeuvre de cette loi de 2016, ainsi que la portée insuffisante du statut de lanceur d'alerte qu'elle a créé, tant du point de vue de la protection contre les représailles que de l'efficacité des dispositifs de recueil et de traitement des alertes.

La commission des lois a certes conservé plusieurs dispositions tout à fait bienvenues du texte adopté par l'Assemblée nationale. C'est le cas de l'extension de la protection à certains tiers exposés ou encore de l'abolition de la hiérarchie entre canaux de signalement internes et externes, rendues nécessaires par la transposition de la directive, qui faciliteront

au renforcement des sanctions civiles, ainsi qu'à la sanction pénale applicable aux représailles. Je pense enfin, s'agissant de l'indispensable accompagnement du lanceur d'alerte, à la faculté, pour les autorités recueillant les signalements externes, d'organiser un soutien financier et psychologique. Notre groupe approuve pleinement ces dispositions. La commission a d'ailleurs amélioré un certain nombre de points dans le texte, en y inscrivant notamment l'obligation pour les autorités externes de rendre compte annuellement de leur action au Défenseur des droits.

Ce faisant, la commission est ainsi revenue sur un apport important de la loi Sapin II, dont elle a minoré l'ambition tout en introduisant une grande complexité pour tous les acteurs. Aussi, nous saluons et soutenons vivement la proposition de notre rapporteure de revenir finalement sur ces modifications et de rétablir la définition de l'Assemblée nationale. Nous présenterons un amendement en ce sens et proposerons d'en tirer les conséquences sur les conditions de la divulgation publique, afin de ne pas restreindre les avancées de la directive à son seul champ.

impose que toutes les personnes qu'elles aident respectent les conditions, notamment de bonne foi, ainsi que les canaux de signalement prévus. Nous proposerons donc de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale,

Verzelen. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, certaines révélations ont entraîné une prise de conscience majeure, au point de modifier notre perception de la réalité. Elles ont parfois conduit à des changements législatifs d'ampleur. Irène Frachon- d'autres l'ont souligné -est probablement l'une des plus emblématiques lanceuses d'alerte françaises de ces dernières années. Depuis, bien des scandales ont éclaté parce qu'une personne a porté à la connaissance du public les abus d'une organisation, d'une entreprise ou d'une association. La valeur ajoutée de ces informations, qui contribuent à alimenter et à faire vivre nos démocraties, est certaine. Internet et les réseaux sociaux ont révolutionné l'accès à l'information. Relais majeurs de l'opinion, ils ont accru l'attente de nos concitoyens en matière de transparence. notre pays fait partie des précurseurs. Depuis l'adoption de la loi Sapin II en 2016, la loi française a d'ailleurs inspiré la loi européenne. Les propositions de loi du député Sylvain que nous examinons aujourd'hui ont notamment pour objectif de transposer les évolutions du droit européen contenues dans la directive du 23 octobre 2019. La loi Sapin II était une avancée notable, mais il est apparu que son dispositif pouvait être perfectionné.

un panel de mesures plus indirectes, visant à rendre la vie impossible à celui qui a osé parler. Les propositions de loi envoient un message clair : les représailles contre les lanceurs d'alerte en raison de leurs révélations sont interdites. Des mesures sont également prévues pour soutenir les lanceurs d'alerte qui en auraient besoin. Les textes rappellent que ce régime de protection n'a vocation à s'appliquer qu'à ceux qui en respectent les procédures établies, ces procédures visent à garantir un équilibre nécessaire entre la protection du secret et la diffusion d'informations d'intérêt général. Les propositions de loi refondent également les modalités de la communication des alertes. Les lanceurs d'alerte devront avertir soit leur organisation en interne, soit une autorité externe désignée par décret. Si ces notifications restent sans effet, les lanceurs d'alerte pourront alors divulguer les informations au public.

domaines sont en outre exclus du lancement d'alerte : ceux qui intéressent la défense nationale et ceux qui sont couverts par le secret médical ou par le secret de l'avocat. Ces conditions nous semblent nécessaires au respect de l'intérêt général. le régime de protection des lanceurs d'alerte prévu par ces textes est soumis à plusieurs conditions, cela ne signifie pas pour autant que la liberté d'alerter soit restreinte. Chacun conserve la possibilité de dénoncer des faits hors de ce régime de protection. Même s'ils ne sont pas strictement concernés par le texte que nous examinons, je veux ici, comme d'autres, rendre hommage à celles et ceux qui travaillent chaque jour à l'information de nos concitoyens. Les journalistes accomplissent un travail fondamental pour alerter l'opinion. Bien souvent, ce sont à eux que les lanceurs d'alerte s'adressent. C'est à eux qu'il revient ensuite de vérifier les informations, de les recouper et de prendre la responsabilité de les publier ou non. À cet égard, je rappelle à quel point le respect du secret des sources des journalistes est capital pour notre démocratie et pour le respect de nos libertés. Nous devons veiller, évidemment, à les protéger au mieux. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre démocratie a besoin à la fois de secret et de transparence.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les propositions de loi ordinaire et organique que nous examinons ce matin visent visent à renforcer la protection des lanceurs d'alerte amenés à signaler des informations sensibles ou confidentielles dans l'intérêt de la société et étant par là même susceptibles de faire l'objet de mesures de représailles ou de voir leur responsabilité engagée. À ce jour, le statut de lanceur d'alerte en France est très largement façonné par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus communément appelée loi Sapin II. le 9 décembre 2016, cette dernière confère en effet à la notion de lanceur d'alerte sa première définition générale en droit positif français. Elle a également permis de mettre en place une armature juridique davantage encline à protéger les lanceurs d'alerte Dans le prolongement de l'entrée en vigueur de la loi Sapin II, l'Union européenne a adopté une directive, qui vise à imposer un cadre minimal pour la protection des lanceurs d'alerte dans les États membres de l'Union. La mise en application de cette directive implique l'établissement d'un nouveau cadre de protection des lanceurs d'alerte par les États membres. En ce sens, je m'associe bien évidemment au triple objectif qui est porté par ces propositions de loi ordinaire et organique et organique : la consolidation du régime français des lanceurs d'alerte, la transposition en droit français de la directive d'octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et l'articulation de cette directive avec le droit national en vigueur. Nul ne peut nier que le texte de l'Assemblée s'efforce de poser les premiers jalons et d'aménager cette articulation, tout en étendant les mesures de la directive au-delà de son champ initial. Le texte transmis par nos collègues députés contribue dès lors à assouplir de nombreux éléments d'encadrement des lanceurs d'alerte issus de la loi Sapin II. En outre, la proposition de loi organique prévoit plus spécifiquement de conférer un rôle d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte au Défenseur des droits. Bien évidemment, notre commission des lois a accueilli favorablement le renforcement du statut des lanceurs d'alerte prévu par ces deux textes, dans la continuité de l'esprit de la directive de 2019 et des recommandations formulées alors par le Conseil d'État. Souscrivant à ces objectifs, la commission a toutefois veillé, scrupuleusement, me semble-t-il, à parfaire l'équilibre nécessaire entre, d'une part, la protection des lanceurs d'alerte et des personnes qui leur portent assistance et, d'autre part, la sauvegarde des secrets protégés et des intérêts matériels ou moraux des personnes mises en cause. Dans cette optique, notre commission a apporté un certain nombre de compléments et d'améliorations rédactionnelles au texte transmis par l'Assemblée

les travaux de notre rapporteur, que je salue, ont permis de clarifier le champ de l'irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d'alerte pour les informations divulguées, mais également de limiter ce champ aux informations dont la révélation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Notre commission a également adopté un certain nombre de modifications visant à mieux articuler les protections introduites par ce texte avec les différents régimes sectoriels déjà existants dans le code du travail ou dans le code général de la fonction publique.

Permettez-moi, enfin, d'évoquer les dispositions introduites par notre commission, afin de veiller à la protection des lanceurs d'alerte contre les procédures bâillons et autres mesures de représailles. En l'état, l'article 10 permet dorénavant au juge d'ordonner la réaffectation d'un lanceur d'alerte à son poste précédent dans le cas où ce dernier aurait fait l'objet d'un changement d'affectation et non pas uniquement en cas de non-renouvellement, de licenciement ou de révocation, ainsi que le prévoyait le texte transmis La proposition de loi amendée prévoit enfin, conformément à la directive européenne, qu'une personne ayant effectué de mauvaise foi un signalement auprès d'une autorité externe s'expose aux peines prévues en cas de dénonciation calomnieuse. Notre commission a en effet adopté un amendement qui insère un nouvel article 9-1 au sein de la loi Sapin II. Ce dernier réprime le fait d'adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité interne ou externe par les peines prévues à l'article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse. La notion même de mauvaise foi implique, pour rappel, l'intention de nuire et la connaissance, partielle, de l'inexactitude des faits. Une telle disposition me semble particulièrement opportune, à l'heure

Ce texte est assez complexe puisque, par définition, la protection des lanceurs d'alerte se situe à la jonction de beaucoup d'autres domaines du droit. Je tenterai de m'en tenir à l'essentiel. De quoi et de qui parle-t-on ? Dans un monde qui, de fait, est de plus en plus complexe, un monde où l'innovation technique, mais aussi juridique et financière ne cesse de croître, bien souvent, seules les personnes qui travaillent dans certains domaines ont la compétence d'en révéler les failles. à l'intérieur de Facebook, où l'on manie les algorithmes, à l'intérieur de PricewaterhouseCoopers (PwC) où l'on fabrique les montages des rescrits fiscaux, à l'intérieur de la centrale de Tricastin quand on est un expert de la sûreté, là et seulement là que l'on accède à certaines informations, mais surtout que l'on est capable de les décrypter. Protéger les lanceurs d'alerte, c'est donc bien sûr protéger des individus qui, du fait de la nature de leurs actions, se mettent très souvent dans une situation d'extrême vulnérabilité, mais c'est aussi protéger l'État de droit.

Très souvent, les lanceurs d'alerte révèlent des faits qui ne sont pas illégaux au moment où ils les dénoncent. Très souvent, les dénonciations précèdent l'illégalité des faits, car c'est grâce aux révélations que l'on est en mesure de légiférer. Quand Antoine Deltour a révélé les pratiques des rescrits fiscaux permettant légalement à des entreprises d'échapper presque totalement à l'impôt au Luxembourg, légalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est grâce à ses révélations que la Commission européenne a lancé une enquête et a conclu, quelques mois plus tard, que ces rescrits fiscaux étaient illégaux. Il est donc primordial d'en rester à une définition large, qui couvre les révélations concernant un crime ou un délit, bien sûr, mais au-delà, une menace, un risque ou un préjudice pour l'intérêt général.

Peu importe qu'un tiers ait acheté l'information ou non. Peu importe que le lanceur d'alerte révèle des faits parce qu'il s'est disputé avec quelqu'un ou parce qu'il veut impressionner quelqu'un. Ce qui importe, dans la directive européenne et dans les faits, c'est réellement l'information. On se moque totalement des sentiments du lanceur d'alerte. L'information est-elle vraie ? Est-elle d'intérêt général ? Telles sont les seules questions qui doivent nous intéresser juridiquement.

d'autres voient en eux des activistes radicaux surpolitisés, qui souhaitent détruire le capitalisme, les entreprises ou se venger de leur supérieur hiérarchique pour de très mauvaises raisons.

C'est pourquoi il faut leur permettre de divulguer les informations publiquement quand cela est nécessaire, ce que personne ne fait de bon gré. Le lien avec le régime d'autres secrets protégés par la loi

Bocquet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique, soulevant la question des droits fondamentaux que sont la liberté d'expression d'une part et la liberté d'information d'autre part. Au-delà de la portée du signalement se pose la question des conséquences auxquelles nos concitoyens et concitoyennes s'exposent en lançant l'alerte et donc de la protection que la société doit leur apporter. Si la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a marqué certains progrès dans la protection des lanceurs d'alerte, elle doit, à l'occasion de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019, être renforcée afin de tirer toutes les conséquences de l'évolution du droit et des travaux européens.

sur les points suivants : la définition étendue des lanceurs d'alerte, la clarification des canaux internes et externes permettant de lancer l'alerte, le renforcement sensible de la protection des lanceurs d'alerte et des sanctions pénales et/ou civiles civiles contre les responsables de procédures abusives ou encore la meilleure reconnaissance des facilitateurs, qui accompagnent les lanceurs d'alerte

Ainsi la commission des lois a-t-elle initialement modifié la définition des lanceurs d'alerte, en supprimant la notion de « menace ou de préjudice pour l'intérêt général ». Cette modification était d'une particulière gravité, car elle visait à remettre en cause l'avancée démocratique la plus forte de la loi Sapin II, qui prévoyait la protection des lanceurs d'alerte non seulement lorsqu'ils dénoncent une violation de la loi dans un cadre professionnel, mais aussi quand ils relèvent un fait qui constitue un préjudice pour l'intérêt général. La proposition de loi Waserman étendait cette définition en supprimant la notion ambiguë de désintéressement.

Avec une telle définition des lanceurs d'alerte, Antoine Deltour, qui a révélé l'optimisation fiscale agressive des multinationales dans le cadre des se serait vu refuser toute protection.

aux chercheurs qui ont révélé depuis plus de vingt ans les effets nocifs des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur les insectes pollinisateurs. » Pourtant, nous le savons, nos concitoyens sont demandeurs d'une plus grande transparence sur tous ces sujets. Dans le monde nouveau dans lequel nous vivons, la lutte contre ceux qui portent atteinte à l'intérêt général est non plus l'apanage de certains, mais bien le droit de tous et de toutes. Pour toutes ces raisons, et malgré les quelques bonnes mesures introduites par la commission des lois, nous voterons contre la proposition de loi en l'état, en comptant beaucoup sur le débat et sur les contributions des uns et des autres pour restaurer et améliorer le texte de l'Assemblée nationale. En parallèle, En parallèle, nous voterons pour la proposition de loi organique, qui permettra l'accompagnement des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits. Comment notre Sénat, si soucieux de la défense des libertés fondamentales, pourrait-il voter un texte de régression ? Mes chers